? ... Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de finances pour 2021, adopté par l'Assemblée nationale

en ce qui concerne la résidence principale durant le quinquennat du président Hollande, mais il est difficilement acceptable que la transmission de la propriété familiale soit assujettie au paiement de droits de mutation à titre gratuit dans le cadre d'une succession. En effet, les revenus qui ont permis d'acquérir cette résidence principale ont eux-mêmes déjà fait l'objet de prélèvements fiscaux. Cet amendement s'inspire des travaux du député Julien Aubert, que je salue à cette occasion

Il s'agit d'alléger la fiscalité applicable aux bénéficiaires d'une transmission à titre gratuit de biens ruraux loués par bail à long terme, lorsque les bénéficiaires s'engagent à le conserver plus longtemps. Ainsi, il est proposé de porter l'exonération de

la stabilité du foncier étant indispensable à la pérennité des exploitations. C'est particulièrement vrai pour les exploitations viticoles, mais cela vaut aussi pour d'autres types de de culture et de foncier. Pour favoriser cette stabilité, je propose d'alléger la fiscalité applicable aux bénéficiaires d'une transmission à titre gratuit de biens ruraux loués par bail à long terme, j'y insiste, lorsque ses bénéficiaires s'engagent à les conserver plus longtemps. Aujourd'hui, l'exonération de 75 % s'applique à concurrence de 300 000 euros si les bénéficiaires conservent les biens reçus pendant au moins cinq elle est ramenée à 50 % au-delà de cette limite. Je propose d'appliquer l'exonération de 75 % jusqu'au double de ce plafond, soit 600 000 euros, lorsque les bénéficiaires s'engagent à doubler la période de conservation, soit dix ans au lieu de cinq ans. Je précise qu'avec cette durée de dix ans l'engagement pris ne ferait pas obstacle à une nouvelle transmission à titre gratuit, puisque, dans ce cas, l'engagement de conservation serait transmis à l'ayant cause.

Je veux d'abord rappeler aux différents auteurs de ces amendements que les conditions de transmission ont déjà été notablement améliorées lors de la loi de finances 2019, avec la revalorisation importante du plafond de déduction à 75 %. C'est d'ailleurs plus avantageux dans le champ agricole que dans bien d'autres secteurs.

plus en plus longues, peut se retourner contre les bénéficiaires, qui, parfois, peuvent se retrouver bloqués. Ensuite, je me dois de signaler que ces ces mesures se heurtent à un problème de constitutionnalité, puisque le Conseil constitutionnel tend à apprécier ces exonérations à l'aune des engagements personnels du bénéficiaire, la simple conservation des biens n'étant pas équivalente à un engagement d'exploitation personnelle. J'émets donc un avis de sagesse.

tout en assurant la paix des familles, et de faciliter les transmissions de patrimoine aux jeunes générations. Il tend ainsi à exonérer ces opérations de tout droit de

après l'article 789 du code général des impôts, afin d'étendre aux legs consentis aux petits-enfants l'abattement

parce que l'intégration des donations réalisées il y a plus de quinze ans à une donation-partage bénéficie déjà d'un traitement fiscal

de taxe de publicité foncière constitue dans le même temps une perte de recettes pour les collectivités territoriales. Je demande également le retrait de l'amendement n° I-473 rectifié. Il y a bien une asymétrie entre les régimes fiscaux des donations et des successions au profit des petits-enfants, une asymétrie qui vise justement à encourager la circulation du capital entre les générations, mais en privilégiant les donations du vivant.

sur le donateur. Il faut ainsi avoir moins de 80 ans pour bénéficier de ce régime de faveur. Il nous semble que cette limite d'âge ne tient pas compte de l'augmentation

car je pense que la limitation de l'âge à 80 ans est peut-être d'abord et surtout une mesure anti-abus. Il s'agit d'éviter que les dons de sommes d'argent consentis en franchise d'impôt

pour tous ceux qui ont dépassé la vingtaine d'années aujourd'hui dans notre assemblée, et puis aussi pour ceux qui, comme moi, commencent à prendre un peu de recul sur l'existence. Entre 90 ans et 100 ans, il se passe tout de même dix ans. Il faut penser aux enfants, ces « bambins » de 70 ans ou 65 ans qui viennent de prendre leur retraite et qui ont besoin de faire face

Cependant, cette somme est forfaitairement estimée à 1 500 euros sans justificatifs, ce qui ne correspond absolument pas au cours du marché actuel, puisqu'elle fait référence à une loi du 30 décembre 2002, qui n'a jamais été actualisée.

quand même le simple cours de l'inflation ou des revalorisations indiciaires. Je rappelle que le dispositif de votre amendement est finalement une tolérance légale,

pas pour objet de compenser le coût exact des frais d'obsèques, et, comme parfois dans d'autres domaines, on pourrait craindre qu'il n'y ait, de ce fait,

», afin qu'une exonération de l'impôt de mutation par décès lors des successions, une exonération des droits de mutation pour les dons en numéraires, ainsi qu'un dégrèvement de la taxe d'habitation, de la contribution à l'audiovisuel public et une décharge de paiement des cotisations de l'impôt sur le revenu restant dues à la date du décès leur soient appliqués,

de guerre ». Je ne suis pas particulièrement convaincu qu'il faille aller jusque-là, mais je vais solliciter, en priorité, l'avis du Gouvernement,

l'avis du Gouvernement ? Le Gouvernement privilégie d'autres voies, d'autres moyens pour reconnaître l'engagement des soignants, notamment la reconnaissance de la maladie professionnelle, mais aussi l'accompagnement des enfants lorsqu'il y a malheureusement eu décès. Nous considérons, comme M. le rapporteur général, que l'exonération de droits de mutation et de fiscalité conduirait à une rupture du principe d'égalité. Par ailleurs, votre amendement, en tout cas celui que vous défendez comme amendement de repli, amènerait à n'en pas douter énormément de demandes reconventionnelles. C'est un avis défavorable pour ces seules raisons. Il s'agit non pas de nier, j'y insiste, l'engagement de ceux que vous visez par l'amendement, mais de privilégier d'autres moyens pour les accompagner et les soutenir.

M. Julien Bargeton. Cet amendement de notre collègue Didier Rambaud vise à étendre aux fondations d'utilité publique la possibilité de recevoir des dons meubles de la part de l'État ou des organismes d'État. Aujourd'hui, cette possibilité vaut pour les associations d'utilité publique, mais n'a pas été étendue aux fondations d'utilité publique. C'est ce que vise cet amendement, avec les mêmes règles de seuil et les mêmes conditions, c'est-à-dire

8 . L'amendement n° I-61, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, C'est un amendement de suppression de l'article. En fait, il n'y a pas de désaccord sur le fond de l'article, mais, pour des considérations techniques, nous proposons qu'il soit examiné en seconde partie.

dotations et que l'éventuelle plus-value réalisée ne soit imposée qu'au moment de la cession future des titres transmis par la fondation bénéficiaire de la transmission. cela tend à garantir la neutralité des opérations de transmission à la date de leur réalisation, sans pour autant aboutir à une perte de recettes fiscales dans le cas où les titres seraient cédés par la FRUP.

créé par la loi Pacte, constitue en fait un nouveau modèle de fondation d'actionnaires, puisqu'il reçoit à titre gratuit des titres ou actions d'une société et tire ses ressources de ces titres. Depuis la loi de finances pour 2020, l'apport de titres au fonds de pérennité est traité comme une opération intercalaire, ce qui signifie que l'imposition des plus-values est reportée jusqu'à la cession future des titres transmis. Je demande l'avis du Gouvernement sur la pertinence de ces amendements, étant donné que la fondation reconnue d'utilité publique et le fonds de pérennité ont des objectifs bien distincts.

tendent à neutraliser les frottements fiscaux susceptibles d'intervenir lors des transmissions à des fondations reconnues d'utilité publique de titres de société, et ce en cohérence avec la loi Pacte.

est ainsi libellé : La parole est à M. Bernard Buis. L'article 9 prévoit que les éléments accessoires d'une offre composite doivent se voir appliquer le même régime de TVA que les éléments principaux de cette opération. Or il ne fournit pas une définition juridique de la notion d'éléments accessoires dans l'offre composite au regard de la TVA.

de vote. Ce débat avec le Gouvernement pose tout de même le problème de la relation entre une jurisprudence stabilisée et la loi. Si le législateur, notamment du point de vue de l'accessibilité du droit et de la clarté pour l'ensemble des usagers du droit, considère qu'il faut figer et rendre pérenne cette définition de l'élément accessoire de la TVA, qui est tout de même un sujet qui importe à quelques milliers d'acteurs économiques, il me semble, quels que soient les mérites de la doctrine administrative, que cet ensemble de règles a bien sa place dans le code général des impôts.

La directive du 28 novembre 2006 ne prévoit ainsi qu'un taux normal, qui ne peut être inférieur à 15 %, et deux taux réduits. Au-dessus de 15 %, la directive ne prévoit donc qu'un seul taux, le taux normal ; un taux majoré de 33,33 % est donc mécaniquement exclu. Néanmoins il serait possible d'imaginer un droit d'accise, c'est-à-dire un impôt indirect où le montant dû est généralement établi en fonction de la quantité. Les cent plus grandes entreprises mondiales de luxe on peut s'en féliciter ! -un chiffre d'affaires total cumulé de 247 milliards de dollars sur l'année écoulée, soit un supplément de 30 milliards. Nous proposons donc qu'une taxe particulière soit appliquée à ces produits de luxe, dont le commerce ne

monsieur le ministre,

utilisé par les associations agréées de protection civile dans leurs actions de prévention et de secourisme. Cette exonération existe déjà, mais elle est limitée aux bateaux de sauvetage de l'assistance en mer. Étendre le champ de cette exonération permettrait aux associations de la protection civile de mettre à la disposition des volontaires et des bénévoles

la mutualisation de personnel à but non lucratif, particulièrement le dispositif des groupements d'employeurs. Cet amendement vise à exonérer de TVA les services rendus par les groupements d'employeurs à leurs adhérents

du code général des impôts. Il s'agit là d'une véritable occasion de confirmer le soutien du Sénat au prêt de main-d'oeuvre, comme le prévoit le plan de relance, et particulièrement aux groupements d'employeurs qui organisent et sécurisent ce prêt de main-d'oeuvre. Le changement du régime de TVA fait partie des évolutions indispensables d'employeurs. Lorsqu'un groupement intervient à la fois auprès d'associations ou de structures non soumises à la TVA et auprès d'adhérents soumis à la TVA, il est lui-même soumis à la TVA sur l'intégralité des mises à disposition. La facturation de cette taxe à des structures qui ne peuvent la récupérer constitue un frein considérable â l'adhésion de structures de tous secteurs. Cela empêche ainsi de compléter le temps de travail de nombreux salariés, et oblige à la création de groupements d'employeurs à destination exclusive d'adhérents non soumis à la TVA. On considère que l'entrée en vigueur de cette mixité permettrait non seulement de sécuriser les 20 000 emplois existants dans les 2 000 groupements d'employeurs non agricoles, mais aussi de créer environ 10 000 emplois supplémentaires, notamment par la mutualisation d'emplois qualifiés nécessaires aux associations, mais aussi aux collectivités territoriales. Il faut noter que cette possibilité de mixité n'entraînerait pas de perte de recettes pour l'État. Nous pouvons même envisager un développement de ces recettes du fait du développement de l'emploi partagé. En effet, ce sont essentiellement les 1 000 groupements d'employeurs associatifs actuellement non soumis à la TVA qui développeraient leur activité avec des entreprises du secteur marchand soumises à cette taxe. Ces mises à disposition auprès d'entreprises marchandes seraient donc soumises à la TVA. Cette avancée majeure pour le développement des groupements d'employeurs s'accompagnerait de la mise en place d'une comptabilité séparée, qui permettrait de bien distinguer les mises à disposition soumises à la TVA de celles qui

dès lors que le pourcentage des recettes donnant lieu au paiement de la taxe est inférieur, pour chacun des membres pris individuellement, à 20 % de leurs recettes totales. Par ailleurs, un groupement peut rendre des services à des personnes non membres assujetties à la TVA, sous réserve que ces prestations soient soumises à cette taxe au taux applicable aux services concernés et

l'ensemble des partenaires sociaux de la branche du sport ont fait le choix d'un nouvel opérateur de compétence, l'Afdas. Les associations employeuses doivent désormais verser une cotisation de formation à ce nouvel opérateur, ce qui a malheureusement eu des conséquences

en raison de leur statut associatif, récupérer la TVA. Cet amendement vise donc à exonérer les petites associations sportives de la TVA sur les opérations de formation pour leurs dirigeants bénévoles et leurs salariés ; le

Le Gouvernement promet depuis des mois la publication d'une stratégie nationale de déploiement des solutions de biocontrôle. L'application d'un taux de TVA de 20 % à la vente des macro-organismes, ainsi que des produits à base de phéromones utilisés en biocontrôle sous forme de piégeage de surveillance, apparaît donc des plus contradictoires avec cette volonté affichée. Cet amendement a pour objet de clarifier les taux de TVA applicables aux produits de biocontrôle. proposons d'inscrire clairement dans le code général des impôts que l'ensemble de ces solutions bénéficient du taux intermédiaire de 10 %. En effet, pour soutenir réellement la transition agroécologique

Cet amendement vise à appliquer un taux de TVA réduit de 2,10 % aux produits issus de l'agriculture biologique, transformés et non transformés. Ce taux est aujourd'hui appliqué aux médicaments.

Je pense qu'il est temps d'avoir une action déterminée en faveur de la démocratisation de ces produits, qui sont- on le sait maintenant, c'est absolument démontré -bénéfiques pour la santé, en termes de prévention.

Je ne vais pas entrer dans le fond du débat, dans la mesure où notre alimentation est suffisamment diverse. Je pense qu'il faut être attentif à tous les produits élaborés

lors que l'on a des produits de qualité, la diversité est aussi importante ; c'est d'ailleurs le choix de nos concitoyens.

invoquée sur tous les sujets. Lorsque l'on souhaite créer des taux nouveaux, c'est irrecevable ! Lorsque l'on veut faire des transferts de listes à l'intérieur des taux, c'est irrecevable ! Mais on ne sait pas pourquoi c'est irrecevable.

n'est donc plus dans la loi de finances que se gère aujourd'hui la TVA. On peut le regretter, mais là, on se fait plaisir : cela fait déjà deux ou trois ans que je regarde tous ces amendements avec une grande circonspection. Nous qui faisons la

débourrés ? Cet amendement vise à appliquer le taux de TVA de 5,5 % aux équidés d'élevage pendant les dix-huit premiers mois de leur vie,

et rédigé avec l'appui de l'inspection générale des finances, indique : « Avant sa troisième année, un cheval de selle sans disposition pour le sport, pourra en effet être destiné à la filière bouchère. De la même manière, la destination d'un cheval de course n'est pas déterminée avant l'âge de 3 ans, qui correspond à son entrée dans le circuit d'entraînement et de sélection des chevaux de course. »

J'ajoute que ces activités d'élevage sont souvent assurées par des agriculteurs, qui en font une forme de diversification leur permettant d'assurer la viabilité de leur exploitation.

est ainsi beaucoup plus général, comprenant les équidés jusqu'à 4 ans, à l'exception de ceux dont la destination a été déterminée plus tôt par leurs premières mises en course ou en compétition, et qui sont normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires

Mme Loisier a eu raison de souligner qu'un travail de redéfinition et de révision de la doctrine était ouvert. Je souhaite qu'il permette de trouver quelques marges de manoeuvre, sans revenir sur l'objectif d'intégration et d'harmonisation ; le défi n'est pas très facile à relever.

Plusieurs des amendements proposés par M. Vogel présentent les risques habituels en matière de TVA, notamment quant à leur acceptabilité. Nous avons travaillé sur la rédaction et sur la formulation proposées par Mme Loisier à l'amendement

style de débat en public. Les ? Non, je vais le retirer, madame la présidente. Je pense, mes chers collègues, que, comme toujours, le mieux est l'ennemi du bien, et que si nous abordons ce sujet avec un spectre trop large, nous risquons, ainsi que l'a dit M. le ministre, de ne pas passer le filtre européen. Je vous invite donc à essayer d'optimiser la démarche que nous avons réussi à mettre en place et qui pourrait aboutir. Le terme de « poulain » est volontairement générique. Il sera précisé

dont, en général, dans nos assemblées- au Sénat particulièrement -, on privilégie le travail collectif, notamment avec les parlementaires concernés et investis sur un certain nombre de sujets.

à l'instant les réserves exprimées sur ce point eu égard à nos engagements communautaires - constitue l'instrument pour atteindre cet objectif. L'idée est de favoriser la réparation des biens et leur reconditionnement. Cela concerne en particulier les biens électroniques et les biens électroménagers, mais pas seulement : c'est la raison pour laquelle il est proposé que ces biens, lorsqu'ils font l'objet de réparations ou de reconditionnements, se voient appliquer un taux de TVA de 5,5 %. C'est une manière de 5,5 %. C'est une manière de nous inscrire dans l'accompagnement des transitions et dans la lutte contre le réchauffement climatique. L'amendement

incorporant au moins 80 % de matières recyclées, afin d'encourager une gestion durable de nos ressources. L'amendement n° I-875 rectifié, présenté par

elle vise les activités liées à la réparation et au réemploi, ce qui permet d'allonger la durée de vie de produits, tout en créant des emplois non délocalisables.

Alors que les derniers mois ont permis un essor considérable de la pratique du vélo, il est urgent d'encourager les Français à pratiquer cette activité physique. Le savoir-rouler est d'ailleurs devenu depuis quelques mois un savoir fondamental inscrit dans le code de l'éducation. Alors que de nombreux Français possèdent un tel équipement, l'abaissement du taux de TVA sera un soutien supplémentaire pour sa remise en état, en plus du « coup de pouce vélo » qui a fait ses preuves, mais qui n'est pas amené à être pérennisé. Cet amendement a été adopté par les députés avant de faire l'objet d'une seconde délibération à la demande du Gouvernement et d'être rejeté.

vise à appliquer un taux de TVA à 5,5 % sur les produits et matériaux issus de matières premières biosourcées gérées durablement. Une étude publiée par l'Ademe au mois d'octobre 2010 conclut que la dépense fiscale induite par la baisse de la TVA serait compensée par la diminution des coûts publics en matière de pollution, santé et ressources.

dont le bois, que ce soit pour la construction ou la rénovation. Je parle à l'imparfait, car, cet amendement étant contraire aux règles de l'Union européenne, nous allons commettre un hara-kiri politique en le retirant.

Il me semble donc possible d'étendre cette possibilité aux travaux de rénovation utilisant des matériaux vertueux et favorisant les filières et les compétences locales. Nous ne connaissons pas, à ce stade, le coût du dispositif,

Cette mesure se fixe un double objectif : accélérer la transition écologique et soutenir notre filière bois, qui est vitale dans nombre de nos territoires et qui permet de promouvoir les emplois non délocalisables.

a été adopté par le Sénat lors de l'examen du PLFR 3 au mois de juillet dernier et vise à appliquer le taux réduit de TVA à tout achat de bois labellisé ou certifié attestant de son caractère local et durable.

à des bois produits dans nos territoires. Nous limitons ainsi les importations et les intermédiaires pour nous tourner vers les filières de bois locales en provenance de forêts françaises. Nous favorisons aussi une économie durable. Nous incitons nos concitoyens à utiliser des bois provenant de forêts exploitées durablement

également d'accompagner la filière bois et forêts, qui fait face à une double crise : le secteur est affecté par la crise sanitaire et économique liée à la covid-19, les principaux acheteurs, tels que le secteur du BTP, tournant au ralenti. La filière accuse le coup, les communes forestières sont à la peine. À cela s'ajoute la concurrence internationale, qui est souvent moins chère à l'achat, car elle répond à moins d'exigences sociales et environnementales. Cette baisse de la TVA orienterait le consommateur vers ces matériaux biosourcés

et solidaire prévoit que le commerce équitable a pour objet d'assurer le progrès économique et social des travailleurs en situation de désavantage économique, du fait de leur précarité, de leur rémunération et de leur qualification, organisés au sein de structures à la gouvernance démocratique. Les entreprises concernées participent à des actions de sensibilisation à des modes de production et de consommation socialement et écologiquement durables. Il convient donc d'encourager ces produits par rapport aux produits classiques, qui présentent des externalités négatives. À ce titre, cet amendement vise à appliquer un taux réduit de TVA de 5,5

de gaz à effet de serre. Dans le contexte actuel, il semble encore beaucoup plus intéressant de ramener le taux de TVA à 5,5 % pour contribuer au développement des transports en commun, qui sont mis à mal en ces temps de pandémie. La

avant d'être fixé à 10 % en 2014. Une telle baisse de TVA permettrait d'accroître la capacité financière des autorités organisatrices de mobilité, qui pourraient ainsi investir dans les réseaux de transports en commun

L'autopartage permet de passer d'une logique de propriété à une logique d'usage. Ainsi, une baisse de TVA à 5,5 % serait l'expression d'un soutien au développement des mobilités douces et partagées, dans le sens des objectifs définis par la loi

La France dispose d'un des écosystèmes les plus riches s'agissant des nouvelles mobilités : trottinettes électriques, scooters partagés, covoiturage, autopartage ... Une telle mesure permettrait de le renforcer.

billets de train de 10 % à 5,5 %. En effet, le train constitue l'un des moyens essentiels pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et de neutralité carbone à l'horizon 2050. Par ailleurs, une politique tarifaire rendant plus accessible le train

à une baisse très importante de la fréquentation en raison de la crise sanitaire. Je souscris

un vecteur significatif pour orienter le consommateur sur ces nouvelles formes de production de ciment. La parole est à M. Daniel Salmon, pour explication de vote.

pour sauver les secteurs de l'hébergement touristique, des cafés et de la restauration. Comme vous le savez, ces secteurs ont été parmi les plus touchés par les conséquences de la fermeture administrative et du confinement de la population.

Sa survie est désormais en jeu, avec des milliers d'emplois à la clé. Les hôteliers font preuve d'initiative. Je pense par exemple à la transformation de chambres en bureaux équipés adaptés aux normes sanitaires pour les télétravailleurs.

Cet outil de la TVA a été utilisé il y a maintenant plus d'une dizaine d'années, avec un succès très limité sur laquestion du prix et de l'emploi.

moi-même travaillons également sur un dispositif d'accompagnement de la sortie progressive du confinement, dès lors que celle-ci sera possible- je ne préjuge en rien des décisions qui seront annoncées demain.

les billets de spectacle, les manifestations théâtrales, les concerts et les parcs zoologiques. J'espère que cet amendement « interstitiel » recevra l'agrément de notre assemblée.

que n'ont pas les musées privés, notamment en matière d'amplitude des horaires d'ouverture au public, de conservation ou de modalités de gestion. C'est la raison pour laquelle j'émets un avis défavorable

La crise sanitaire a durement frappé l'ensemble du monde de la culture, y compris le secteur des médias. Au sein de notre paysage audiovisuel, les télévisions locales assurent une véritable mission de service public et couvrent 70 % de la population française. En diffusant des des informations de proximité, ces chaînes locales valorisent les acteurs économiques, sportifs, sociaux et culturels du territoire. Leurs moyens de fonctionnement reposent à la fois sur des recettes privées et le soutien des collectivités locales. Sur un marché qui s'est quelque peu autorégulé, seules les plus qualitatives et celles qui sont dotées d'un modèle économique viable subsistent. Dans le contexte actuel, le budget des chaînes locales risque d'être fragilisé. Cet amendement vise donc à leur apporter une aide sous la forme d'un taux réduit de TVA applicable aux dotations versées par les collectivités.

de la crise, comme l'ensemble de la presse, mais elles ne bénéficient ni des recettes publicitaires ni des aides directes et indirectes de l'État. Cet amendement a déjà été adopté par le Sénat, sur l'initiative de David Assouline, il y a deux ans, lors de l'examen du PLF pour 2019. Cette disposition n'a pas été retenue dans la suite de la discussion budgétaire, mais il me semble que la crise de la presse et les conditions dans lesquelles exercent les agences de presse méritent toute notre attention

prévoit une baisse du taux de la TVA à 5,5 % sur les ventes de CD, vinyles et téléchargements à l'horizon de 2023, ce délai devant permettre à la France d'emporter l'adhésion des autres États membres sur la modification TVA actuellement en discussion. L'objectif est de préserver le réseau de distribution émaillant l'ensemble du territoire, avec un double enjeu d'accès à la culture et de diversité.

monsieur le ministre, conforter mon avis sur le monopole des lois de finances en matière de fiscalité. En matière de TVA, la définition du terme « sport » est encadrée par les différentes réglementations que nous avons évoquées, qui retiennent

Je confirme le pressentiment de notre collègue Jean-François Rapin : avis défavorable sur ces deux amendements.

européen énoncées par la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 ou par le règlement du 5 avril 2017 qui la remplace. Ces dispositifs comprennent les tests d'acide nucléique (PCR) réalisés par prélèvement nasopharyngé, les tests antigéniques réalisés par prélèvement nasopharyngé et les tests de détection d'anticorps effectués sur un échantillon sanguin. Cette mesure exceptionnelle et temporaire devrait perdurer jusqu'à la fin de la crise sanitaire de la covid-19. Elle ne devrait pas s'appliquer au-delà du 31 décembre 2022.

jusqu'à 150 euros par mois, soit 14 % du budget de 80 % des retraités percevant moins de 1 000 euros par mois. Lorsque ces derniers n'ont pas les moyens de s'en procurer, il peut en résulter des risques graves d'infection avec des conséquences psychologiques importantes conduisant notamment à la désocialisation.

relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée permet aux États membres d'appliquer un taux réduit sur ces produits, comme le font d'ailleurs déjà la Belgique ou les Pays-Bas. La représentation en France de la Commission européenne nous a récemment confirmé que cette directive permettait d'appliquer un taux réduit

que la prévision de croissance pour 2020, à savoir une récession de 11 %, est considérée comme prudente, et que la prévision de croissance pour 2021, eu égard aux chiffres de 2020 et aux conditions de levée progressive de l'état d'urgence sanitaire, est considérée par le Haut Conseil comme cohérente. J'aurai l'occasion de revenir plus longuement sur la nature de cet avis, dont je vous transmets uniquement les éléments les plus succincts, tels qu'ils m'ont été communiqués à l'instant. Cela signifie que, conformément à l'engagement pris jeudi après-midi lors de la discussion générale, j'aurai, lors de la seconde délibération visant à tirer les conséquences des votes du Sénat sur la première partie, l'occasion de vous proposer de réviser l'article